deux semaines, une période de confinement. Je tiens à saluer le civisme de nos compatriotes, qui savent que cette épreuve permettra à tous nos soignants de sauver des vies.

cet hommage. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Paul Natali, qui fut sénateur de la Haute-Corse de 1998 à 2005. Monsieur le Premier ministre, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, il n'avait jamais été sénateur, mais il a siégé au banc du Gouvernement dans notre assemblée.

la crise financière. Nous avions été ensemble au Gouvernement sous l'autorité du président Jacques Chirac. C'était un gaulliste convaincu, un homme cultivé, ayant son franc-parler, dévoué à son pays, à son département et à la ville qui l'avait élu maire en 1983-

Je vous remercie,

du groupe Union Centriste, concerne La Poste. Le groupe La Poste vient d'annoncer « se recentrer sur ses missions essentielles ». En conséquence, depuis lundi, le courrier n'est plus distribué que trois jours par semaine. De plus, La Poste ne maintient que 6 % de ses bureaux ouverts, en horaires aménagés, au cas par cas. Enfin, de nombreux distributeurs de billets de La Banque postale ne sont pas approvisionnés. Les conséquences de ce qui ressemble à une démission sont graves. En milieu rural, certaines personnes se retrouvent totalement isolées. La distribution du courrier trois jours sur six fragilisera un peu plus la presse écrite, sans parler du lien social et d'information qu'elle assure auprès des personnes âgées. Une telle situation est bien peu compatible avec l'idée que les Français se faisaient de ce service public et d'une entreprise qui communique sur sa proximité et son lien avec les territoires. Encore plus grave, cette situation va couper les vivres à certains de nos concitoyens. J'ai été interpellée par une personne âgée ayant pour seule ressource l'argent qu'elle retire au guichet de La Poste. C'est aussi le cas des plus de 1,5 million d'allocataires des minima sociaux, qui viennent chaque mois retirer des espèces. Pour répondre à cette urgence, La Banque postale permettra les retraits d'espèces aux distributeurs à partir du 4 avril, au lieu du 7, et 250 bureaux de poste supplémentaires seront ouverts pour faciliter les retraits aux guichets.

À l'heure où les gens n'ont plus d'argent, où les commerçants commencent à consentir des ardoises, ne peut-on correctement protéger les agents de La Poste afin que le service soit rendu normalement ? Pourquoi seraient-ils plus exposés dans les bureaux que les commerçants de bouche, qui sont ouverts ? N'est-il pas possible, au moins en zone rurale,

assureront le paiement des prestations sociales, afin que tout se passe dans de bonnes conditions. La caisse d'allocations familiales anticipera le versement de ces prestations

en particulier aux plus vulnérables. Le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation. Le Premier ministre m'indiquait à l'instant qu'il ferait le point cette semaine avec les dirigeants de La Poste, pour veiller à ce qu'un

La pandémie que nous subissons met chaque jour en évidence le travail et l'abnégation de tout le personnel soignant qui est en première ligne, mais aussi l'indispensable travail de toutes les personnes qui agissent au quotidien, souvent dans l'ombre, pour faire fonctionner une grande part de notre économie. À toutes ces femmes et à tous ces hommes, je veux dire merci. Pour sortir de cette crise, pour protéger les autres, nous demandons à chacun de se confiner. À tous ces Français qui acceptent l'attente, nous devons aussi dire merci. Nombre de ces citoyens s'unissent et inventent des solutions à des problématiques touchant les plus démunis, les plus vulnérables,

Elle doit permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de donner de leur temps. Cet espace d'engagement a été construit en lien avec les associations humanitaires et aux côtés des collectivités publiques et de leurs structures. Il doit leur permettre de faire état de leurs besoins de renforts dans quatre domaines principaux l'aide alimentaire et l'aide d'urgence, la garde exceptionnelle d'enfants, le lien avec les personnes fragiles isolées et la solidarité de proximité. Monsieur le secrétaire d'État, combien combien de nouveaux bénévoles avez-vous enregistrés sur cette plateforme depuis son lancement ? À titre personnel, je connais des jeunes qui souhaitent prêter main-forte, mais ne trouvent pas de missions dans leur commune. Comment peuvent-ils être utiles ? ? Enfin, quelles missions auront les préfets ? Seront-ils les traits d'union entre l'offre et la demande ? Inciteront-ils les associations à saisir leurs offres de missions ? La parole

250 000 Français ont rejoint la réserve civique pour venir en aide sur le terrain aux plus démunis, et 50 000 d'entre eux sont déjà engagés dans des missions.

mais le risque d'une grave crise économique est devant nous. Le Gouvernement en est totalement conscient et a réagi très rapidement, avec un premier train de mesures consistantes et pertinentes. Le dispositif mis en place mériterait cependant d'être amplifié, complété et parfois précisé.

Ma seconde question porte sur le fonds de solidarité d'un milliard d'euros, qui sera majoré de 200 millions d'euros par les compagnies d'assurance. Du fait de la crise sanitaire et des mesures de confinement, qui entraînent un fort ralentissement des activités, tant économiques que des particuliers,

Ne doit-on pas aller vers la mise en place d'un fonds de solidarité beaucoup plus ambitieux, qui pourrait prendre en charge, même de manière très partielle, les pertes d'exploitation des entreprises et les pertes de revenus des indépendants, artisans, commerçants et professions libérales ?

vous avez raison de souligner l'importance du plan qui a été mis en oeuvre par l'État pour accompagner les entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles. Ce plan repose sur quatre piliers : le chômage partiel, le report des cotisations sociales et fiscales, le fonds de solidarité et la possibilité d'obtenir des financements bancaires garantis par l'État à hauteur de 90 %.

pour financer les commandes de médicaments, de respirateurs et de masques produits chez nous par nos entreprises. Il était temps ! Masques, blouses et gants arrivent au compte-gouttes, il faut bien le dire, et désormais les médicaments, dont le curare, commencent à manquer.

Que dire de celles et de ceux qui travaillent alors que leur activité n'est pas nécessaire en ce moment ? Quand allez-vous réquisitionner les entreprises pour qu'elles fabriquent les médicaments nécessaires, tels le curare ou la morphine, et l'oxygène ? Quand allez-vous engager les moyens nécessaires

autant de respirateurs que la France en a produits en trois ans. Tels sont les faits ! Ces mesures permettent d'accompagner la montée en puissance de nos soignants, que je veux ici remercier pour leur travail remarquable

demain, il vous faudra rendre des comptes aux soignants, mais aussi à la population tout entière. Il faut changer de logiciel, madame la secrétaire d'État ! L'urgence vitale exige de substituer à vos dérives libérales le choix de l'intérêt général. Les réquisitions et les nationalisations sont la voie du bon sens, la voie du salut

sur les plans tant sanitaire qu'économique. Les mesures prises pour freiner puis stopper la propagation du virus sont prioritaires et nécessaires, mais elles frappent aussi très durement nos entreprises et leurs salariés. Qu'elles aient arrêté ou réduit leur activité, celles-ci subissent toutes d'importantes pertes d'exploitation, mettant en question leur survie même. Le Gouvernement a pris des dispositions exceptionnelles pour endiguer cette catastrophe économique et sociale ; elles sont les bienvenues.

modifier, au nom de l'urgence, le code des assurances et déclarer un état de catastrophe naturelle et sanitaire, en élargissant l'indemnisation aux pertes d'exploitation sans dommage aux biens matériels ? Comptez-vous invoquer un motif d'intérêt général impérieux et saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il reconnaisse la validité d'une loi loi rétroactive au premier jour du confinement

étant, puisque vous considérez que ce n'est pas possible, peut-être pourriez-vous envisager une contribution spéciale temporaire des compagnies d'assurance, comme en 2017, de telle sorte que celles qui collectent 2,1 milliards d'euros par an au titre de la couverture du risque de perte d'exploitation aillent au-delà des 200 millions d'euros que vous avez évoqués.

Dans cette crise, les soignants sont en première ligne. Je tiens à saluer leur professionnalisme et leur dévouement. Je tiens aussi à saluer, comme vous l'avez fait, monsieur le président, tous nos concitoyens qui respectent les consignes et restent confinés chez eux ; ils contribuent également à endiguer l'épidémie. Au-delà, je veux saluer les Français qui continuent de remplir leur mission ; je pense aux caissières, aux policiers, aux militaires, aux éboueurs, aux fonctionnaires, aux routiers, aux agriculteurs, à tous ces professionnels qui continuent à travailler malgré les conditions dégradées. Pour mener la guerre contre le virus, notre pays a besoin que chacun soit à son poste. La continuité des services est indispensable au fonctionnement de notre pays cela vaut particulièrement pour nos services publics. Je partage à cet égard l'attachement à la continuité du service postal dans nos territoires ruraux qu'a exprimé Mme Guidez. Il n'est pas acceptable que des bureaux de poste ferment ou que le courrier et la presse ne soient plus distribués ; ce sont souvent, aujourd'hui, les seuls liens avec l'extérieur, notamment pour les plus âgés. L'heure est à la mobilisation générale. La France a besoin, je le répète, que chacun soit à son poste, pour que tout le monde puisse se nourrir, se chauffer, s'éclairer. L'unité nationale est le geste barrière de nos institutions. secrétaire d'État, pouvez-vous nous assurer que, dans les semaines qui viennent, la continuité des services indispensables à la population sera assurée ? J'évoquerai un sujet plus précis, qui tient à coeur à l'Angevin que je suis. Pour assurer la continuité alimentaire, encore faut-il qu'il y ait des producteurs.

à préciser très exactement les conditions dans lesquelles les activités doivent être exercées, à rappeler comment les gestes barrières et les mesures de distanciation peuvent être

accompagner ces mesures. Nous y travaillons également en mettant à disposition, sur une plateforme gérée par la direction générale des entreprises, un certain nombre de matériels de protection pouvant

nous savons tous que la priorité, aujourd'hui, est la sécurité sanitaire et la santé de nos concitoyens. Malgré tout, plusieurs sujets d'ordre économique doivent être rapidement appréhendés.

Le deuxième sujet a trait à la situation économique des petits commerçants. La crise qu'ils traversent les expose de plus en plus au risque de faillite. Alors qu'on leur demande de fermer boutique au motif que leur activité n'est pas jugée prioritaire, les grandes surfaces continuent de vendre des produits qui ne relèvent pas des besoins primaires. des géants du e-commerce, tels qu'Amazon, pour qui la crise constitue une aubaine économique sans égale ? La distorsion de concurrence entre commerce numérique et commerce physique, déjà importante, se trouve renforcée.

des professions libérales, qui désespèrent de la situation, d'autant que les contrats d'assurance ne couvrent pas ces pertes. L'État a annoncé 300 milliards d'euros de prêts bancaires garantis : c'est une bonne chose. Madame la secrétaire d'État, pourquoi ne pas confier ne serait-ce que 5 % de ce montant aux compagnies d'assurance en leur demandant de couvrir les pertes d'exploitation des nombreux professionnels en détresse, au titre des catastrophes sanitaires ? Je vous remercie,

que la presse soit distribuée, y compris en début de semaine, et que les services de proximité assurés par La Poste, notamment auprès des plus vulnérables et des personnes âgées,

maintenant déposer leur dossier pour bénéficier d'une première tranche de 1 500 euros, qui sera payée dans les prochains jours. Elle

et la pratique de l'IVG pour les mineures. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ces trois propositions ? La parole

Elle relaye une question écrite que notre collègue Olivier Cadic, sénateur représentant les Français de l'étranger, vous a adressée la semaine dernière, monsieur le ministre des solidarités et de la santé. Depuis, ses inquiétudes n'ont cessé d'être confirmées par son réseau, qui couvre le monde entier. Si 10 000 de nos compatriotes, selon le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, se battent encore pour se faire rapatrier- je leur adresse ici un message de soutien et de solidarité, car ils se trouvent parfois dans des situations très difficiles -, les 120 000 personnes rentrées depuis deux semaines n'ont eu droit à aucune information à leur arrivée en France. Aussi incroyable que cela puisse paraître, aucune mesure spécifique n'encadre le retour des Français sur le territoire national. Aucune mesure de protection n'a été mise en place. Même s'ils arrivent d'un pays à risque, on ne les met pas en quarantaine, comme on avait pourtant commencé à le faire avec les Français revenant de Wuhan, en Chine.

Cette réalité tranche avec les mesures prises par de nombreux pays, où les voyageurs sont interrogés sur leur état de santé et auxquels on recommande de se confiner. Monsieur le ministre, comment se fait-il que des mesures de rapatriement si drastiques à l'origine, pour les Français revenant de Wuhan, aient pu laisser place à un tel laisser-aller dans les aéroports ? Comment justifiez-vous que les Français soient confinés, mais qu'aucune mesure sanitaire n'organise l'accueil de nos rapatriés ?

Monsieur le Premier ministre, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, je veux, au nom du Sénat et en mon nom personnel, rendre un hommage particulier à Jean-Louis Schroedt-Girard, qui a quitté ses fonctions de secrétaire général du Sénat hier, au terme d'une carrière de trente-huit années au service de notre institution. Son départ intervient dans les circonstances si particulières de l'urgence sanitaire à laquelle une grande partie de l'humanité est aujourd'hui confrontée. Je peux témoigner que, jusqu'au bout, Jean-Louis Schroedt-Girard aura été à nos côtés pour piloter l'administration sénatoriale, à laquelle je rends une nouvelle fois hommage pour la réactivité et l'efficacité dont elle a fait preuve pour permettre à notre institution